J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2021 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

avant la crise sanitaire, l'article L. 642-3 du code de commerce était clair : dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure n'étaient admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise, partielle ou totale, de l'entreprise placée en liquidation judiciaire. Ça, c'était avant.

pour garantir le maintien de l'emploi. Ainsi, l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai dernier, prise sur le fondement du du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit qu'une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise en liquidation judiciaire peut, jusqu'au 31 décembre de cette année, être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Cette disposition prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

oui, pour un certain nombre de grands groupes. On pourrait même parler de grandes familles : sixième fortune de France, la famille Mulliez a eu recours immédiatement à cette ordonnance pour deux de ses entreprises,

les entreprises durant la crise sanitaire, une ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

de se porter acquéreurs dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette interdiction s'explique par un souci bien légitime de moralisation de la vie des affaires. Il s'agit d'éviter la fraude aux intérêts des créanciers, c'est-à-dire que le débiteur ou le dirigeant ne conserve directement ou indirectement tout ou partie des actifs de l'entreprise, alors même qu'il se serait délesté du passif. aussi la fraude à l'assurance contre le risque de non-paiement des créances salariales. En revanche, contrairement à ce que l'on entend parfois, cette interdiction n'est pas destinée à protéger les salariés eux-mêmes contre un détournement de la procédure de licenciement, car les formes prévues par le code du travail pour tout licenciement pour motif économique doivent être respectées. Le droit commun prévoit des dérogations à cette interdiction, en faveur des exploitations agricoles, d'abord, des autres entreprises ensuite, sous réserve des conditions suivantes : le tribunal ne peut ordonner leur cession à l'un des dirigeants, un allié ou un proche de ceux-ci ou du débiteur personne physique que sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé et après avis des contrôleurs. Cette dérogation est toutefois peu utilisée. L'assouplissement prévu par l'ordonnance est d'ordre procédural : il permet au débiteur ou à l'administrateur de former lui-même une requête en vue d'une offre de rachat, sans que le ministère public soit tenu de la reprendre à son compte.

Il est toutefois très encadré : outre que le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs, comme le droit commun l'exige, l'ordonnance rend obligatoire la présence à l'audience du ministère public, qui peut y présenter des observations et, le cas échéant, interjeter appel. En outre, comme toujours en matière de procédures collectives, l'appel du parquet est suspensif. Au surplus, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent : l'offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation des emplois et d'apurement du passif. Cet assouplissement a été motivé par deux raisons très pragmatiques, qu'il est difficile de contester. Sur le plan économique, d'abord, on pouvait craindre que les repreneurs potentiels ne soient beaucoup moins nombreux qu'habituellement dans un contexte économique très incertain. de vue moral, ensuite, les dirigeants d'entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n'en portent aucunement la responsabilité : il pouvait donc paraître légitime de leur permettre de présenter plus facilement des offres de reprise. En outre, un examen attentif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont fait un usage prudent de cette possibilité, le plus souvent avec l'assentiment des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Par exemple, dans le cas de la société Camaïeu, le tribunal de commerce de Lille a retenu l'offre présentée par la Financière immobilière bordelaise plutôt que celle d'un consortium dont faisait partie le dirigeant de Camaïeu, en raison principalement de l'opposition du comité social et économique à cette dernière offre et alors même que les administrateurs, les mandataires, les contrôleurs et le parquet plaidaient en faveur de l'offre du consortium.

la proposition de loi n'aurait aucune chance d'entrer en vigueur, faute d'être définitivement adoptée avant cette date ... Au contraire, j'estime que prolonger l'application de cette mesure aurait pu avoir du sens, éventuellement sous une forme modifiée pour dissiper toute crainte d'abus.

notamment parmi les petits commerces, les TPE et les PME, ce dispositif aurait peut-être pu leur être utile. D'ailleurs, les syndicats de salariés que nous avons entendus se sont montrés plus ouverts sur un dispositif ciblé. ciblé. Telle n'est pas l'intention du Gouvernement, d'après ce que le cabinet du garde des sceaux m'a indiqué lors de mes auditions. Je forme le voeu que l'ordonnance ait au moins permis aux acteurs économiques, aux praticiens des procédures collectives et aux parquets d'être désormais pleinement sensibilisés à la nécessité de faciliter les cessions d'entreprise, y compris à leurs dirigeants si cela se révèle opportun, et d'être mieux informés des souplesses prévues par le droit commun. Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, la commission des lois vous recommande de ne pas adopter la présente proposition de loi.

Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le mois de mars dernier, le Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, mobilise des moyens exceptionnels exceptionnels pour protéger nos entreprises et leurs salariés des conséquences économiques de la crise sanitaire. Le « quoi qu'il en coûte », la solidarité et la combativité des Français ont démontré leur efficacité

ou à leurs parents ou alliés de présenter, avec des précautions et des garanties définies par la loi, une offre d'achat partiel ou total de l'entreprise. Avant d'en venir au fond de cette proposition de loi, je formulerai deux remarques. D'abord, il est inscrit très clairement dans l'ordonnance en question que la simplification introduite prendra fin le 31 décembre 2020, soit très exactement

deux mois. Ensuite, je m'interroge sur l'intitulé de cette proposition de loi : « supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan ». « Après avoir organisé son dépôt de bilan échanger avec un très grand nombre d'entreprises, de toutes tailles, et pour avoir eu, dans une vie antérieure, une expérience au sein d'une entreprise et comme investisseur, je puis vous assurer que je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui organisent sciemment leur dépôt de bilan.

Le quotidien des dirigeants et des salariés, dans ce contexte, ce sont l'incertitude et l'angoisse, la peur de voir les efforts d'une vie s'effondrer en quelques jours, malgré des mois de lutte et des nuits sans sommeil. Cette détresse et cette peur, le Gouvernement les entend. Il met tout en oeuvre, quoi qu'il en coûte, pour soutenir celles et ceux qui ne cessent de se battre, chaque jour, pour sauver leur activité le fonds de solidarité, des prêts garantis par l'État, l'activité partielle la plus protectrice d'Europe pour préserver les salariés, des exonérations de charges sociales. Non, madame la sénatrice, les chefs d'entreprise n'organisent pas la faillite de leur entreprise : ils se battent pour la survie de leur activité ! Au reste, nombre d'entre eux sont préoccupés par la protection de leurs salariés.

tous les atouts de notre côté et tous les outils au service des entreprises en difficulté pour leur permettre de passer ce cap. Tel est le contexte dans lequel a été amodié ce dispositif existant de longue date dans le code de commerce.

ou encore, plus modestement, 59 emplois chez le lunettier jurassien L'Amy- soit, dans les deux derniers cas, l'intégralité des emplois. Le dispositif a donc profité à des entreprises de toutes tailles. Ensuite, il s'agissait de répondre à l'urgence, qui ne permettait pas nécessairement à des repreneurs de se porter acquéreurs d'entreprises, compte tenu des délais très courts et des conditions de travail dégradées pour eux. Ainsi, le dépôt de bilan et la reprise de Novares ont eu lieu alors que le premier confinement n'était pas encore levé. Simplifier ne veut pas dire réduire les garanties protectrices. Dans le droit commun, le débiteur ou les dirigeants disposaient déjà de la faculté de reprendre une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, sur réquisitions spéciales du ministère public, par un jugement spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs.

; il peut présenter des observations et, surtout, interjeter appel, avec effet suspensif. Non, il ne s'agit donc pas d'une régression des protections, non plus que d'un effet d'aubaine. Quand un dirigeant voit son entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, il risque de perdre son outil productif face à une offre concurrente

dans cette procédure, le tribunal de commerce de Lille a suivi l'avis du comité social et économique de l'entreprise, donc la voix des salariés, qui s'étaient prononcés en faveur de l'offre concurrente de celle des dirigeants.

le Sénat a relevé : « Du côté de la Chancellerie, l'on a pu observer un certain flottement dans la gestion de la crise en ce qui concerne ces juridictions. Les présidents des tribunaux de commerce n'ont pas été destinataires de la circulaire du 14 mars 2020 relative à l'adaptation de l'activité pénale et civile des juridictions. De premières directives leur ont été adressées par la dépêche du 19 mars 2020 du directeur des affaires civiles et du sceau, qui invitait les tribunaux de commerce à limiter leur activité aux " affaires urgentes " dans le cadre du contentieux général et à la désignation de mandataires en ce qui concerne le traitement des difficultés des entreprises ; les les tribunaux étaient en revanche invités à surseoir à statuer sur les demandes d'ouverture de procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, considérées comme non urgentes- ce qui ne manquait pas de surprendre. Cette dépêche a été abrogée par la circulaire du 30 mars 2020 [ ...]. « Selon les informations fournies aux rapporteurs avant la survenue de l'épidémie, aucun plan de continuité d'activité n'avait été élaboré au sein des tribunaux de commerce, la Chancellerie n'ayant jamais donné d'instructions en ce sens. Cela n'a pas empêché les chefs de juridiction et les greffes d'organiser dans l'urgence les modalités de travail des magistrats [ ...]. » Madame la ministre, vous avez indiqué que le nombre de dépôts de bilan était le plus faible depuis des années. Certes, mais je ne fais pas exactement la même analyse que vous.

retarder les procédures collectives, mais à un moment ou à un autre, face à la réalité, ou à la suite d'autres confinements si la crise sanitaire devait se prolonger, ce que ni vous ni moi ne pouvons prévoir aujourd'hui, il y aura forcément

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure n'étaient admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise, partielle ou totale, de l'entreprise placée en liquidation judiciaire. Ça, c'était avant. pour montrer combien la loi est protectrice en la matière. L'ordonnance du 20 mai 2020, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit qu'une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise en liquidation judiciaire peut, jusqu'au 31 décembre prochain, être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. La requête aux fins de dérogation à l'interdiction pour certaines personnes de présenter une offre de reprise pouvait être faite avant cette ordonnance, mais uniquement

par cette ordonnance et ses conséquences, quelles que soient les considérations qui ont pu présider à sa mise en oeuvre. Je l'en remercie

ont déjà profité de cet effet d'aubaine pour effacer une partie de leurs dettes, faciliter les licenciements des salariés, faire prendre en charge des salaires par l'Unédic puis

Il est incontestableque cette procédure a eu ou peut avoir des effets pervers. En effet, la possibilité ouverte par l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 est avantageuse puisque, en cas de liquidation judiciaire, les indemnités de licenciement sont prises en charge non par l'employeur, mais par le régime de garantie des salaires, l'AGS. Elles s'élèvent alors au montant minimal prévu par la loi. Or lors d'une restructuration classique, le plan de sauvegarde de l'emploi doit faire l'objet de négociations

qui ont récupéré l'entreprise une fois qu'un certain nombre de charges financières ont été endossées par les autorités publiques. Pourtant,

pleinement sensibilisés à la nécessité de faciliter les cessions d'entreprises, y compris à leurs dirigeants si cela se révèle opportun, et qu'ils étaient mieux informés désormais des souplesses prévues par le droit commun.

ait décidé de ne pas proroger cette mesure montre que cette proposition de loi va dans le bon sens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues,

L'objectif est d'éviter la fraude, qu'elle soit aux intérêts des créanciers ou à l'assurance. La proposition de loi qui nous est soumise ce matin a pour objet d'abroger l'article 7 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, qui a temporairement assoupli- jusqu'au 31 décembre 2020 -la procédure permettant aux dirigeants d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ou à leurs parents ou alliés, ou encore à ceux du débiteur lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de présenter une offre de rachat partiel ou total de l'entreprise. Cet assouplissement prévu par l'ordonnance est d'ordre procédural. Il permet au débiteur ou à l'administrateur de former lui-même une requête en vue d'une offre de rachat sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte.

mais l'ordonnance rend également obligatoire la présence du ministère public à l'audience, au cours de laquelle il peut présenter des observations et, le cas échéant, interjeter l'appel. Dans ce cas, l'appel du parquet est suspensif. Enfin, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent : l'offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation des emplois et d'apurement du passif. proposition de loi, cet assouplissement de la procédure de reprise prévu par l'ordonnance du 20 mai 2020 a constitué un effet d'aubaine pour les dirigeants dont la mauvaise foi ou la mauvaise gestion avaient elles-mêmes contribué aux difficultés de leur entreprise. Nous comprenons bien l'émoi que plusieurs affaires très médiatisées ont suscité. Toutefois, nous partageons la position du ministère de la justice, qui considère que cet assouplissement procédural temporaire se justifie par le risque que les repreneurs potentiels soient beaucoup moins nombreux qu'habituellement en cette période, compte tenu du contexte économique très incertain et du fait que les dirigeants d'entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n'en portent aucunement la responsabilité. Aussi, il apparaît légitime de leur permettre de présenter plus facilement des offres de reprise. Par ailleurs, les juridictions ont fait une application prudente de cette possibilité, le plus souvent avec l'accord des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l'ensemble des circonstances de chaque cas.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le tribunal de commerce d'Orléans a scellé en octobre dernier le sort d'Inteva Products France. Ce groupe, filiale d'un équipementier automobile américain, était en redressement judiciaire depuis le La justice a tranché : c'est la maison mère, candidate à sa reprise, qui rachète son entreprise, après avoir organisé son dépôt de bilan pour une transaction fixée à 1,25 million d'euros. Ce rachat lui permet d'abandonner- excusez du peu -169 millions d'euros de créances Dans les faits, ce rachat entraînera la fermeture de l'usine de Saint-Dié-des-Vosges, qui emploie 223 salariés, ainsi que 42 licenciements sur les 160 postes que compte le siège à Sully-sur-Loire, soit 265 licenciements au total. Voilà un exemple assez parlant de ce que permet l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai dernier. Celle-ci facilite la reprise d'une entreprise en redressement judiciaire par son dirigeant et permet un apurement de la dette, le ou les dirigeants se délestant au passage d'une partie des salariés. Auparavant, une réquisition spéciale du parquet était nécessaire pour pouvoir procéder ainsi. Sinon, il fallait respecter un délai minimum de cinq ans. Le Gouvernement a donc procédé à un sérieux assouplissement de la règle initiale.

Ainsi, de grands groupes se sont engouffrés dans la brèche pour restructurer à moindre coût. C'est le cas d'Inteva Products France, mais aussi de l'entreprise Orchestra Prémaman, qui s'est séparée de plusieurs centaines de salariés, l'opération ayant permis à l'équipe dirigeante de poursuivre l'aventure à peu de frais après l'apurement du passif du groupe, estimé à 500 millions d'euros. On peut citer également l'entreprise Alinéa, qui a supprimé près de 1 000 emplois. Permettez-moi

L'entreprise réduit ses effectifs à moindre coût puisque les licenciés sont indemnisés au minimum, sans aucun complément. Et encore une fois, ce sont les salariés qui paient le prix fort.

Assouplir les règles de droit commun pour faciliter les reprises et éviter les faillites serait sans doute bénéfique dans un monde entrepreneurial tout à fait bienveillant, mais dans celui que nous connaissons, où un certain nombre de chefs d'entreprise agissent d'abord en acteurs économiques cyniques, leur rationalité étant tout entière tournée vers l'optimisation des coûts et la recherche du profit, nous savons que cela se fait trop souvent au détriment des droits des salariés. salariés. Cette disposition doit arriver à terme le 31 décembre. Nous saluons le fait que la commission des lois ait choisi de ne pas la proroger, car tel était le risque. Nous serons attentifs à ce qu'elle ne le soit pas par d'autres canaux légistiques dans les mois à venir. Cette proposition de loi aura eu le mérite d'alerter et d'appeler à la vigilance. Nous notons au passage que l'on n'entend ni le Gouvernement ni la majorité sénatoriale se plaindre de l'endettement de l'État On laisse filer la dette publique pour renflouer les comptes de ces entreprises sur le dos du contribuable, selon un mécanisme- hélas classique -de privatisation des profits et de socialisation des pertes. Demain, on viendra nous expliquer que le coût du service public est insoutenable au regard de l'endettement de la Nation

actuelle, l'article L. 642-3 du code de commerce relatif à la cession des entreprises en liquidation judiciaire pose un principe d'interdiction, pour un certain nombre de personnes, dont les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, de présenter une offre de reprise de cette même entreprise. Le même texte prévoit également que le tribunal puisse déroger à cette interdiction et autoriser la cession à l'une des personnes visées sur requête du ministère public et par jugement spécialement motivé. Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises durant la crise sanitaire, une ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de

La présente proposition de loi de notre collègue Sophie Taillé-Polian vise à supprimer l'article 7 de ladite ordonnance au motif qu'elle créerait un effet d'aubaine pour des patrons voyous et leur permettrait ainsi d'organiser un plan social à moindre coût. Le groupe RDPI partage la position de la commission des lois, qui est défavorable à l'adoption de ce texte. J'en profite pour souligner la qualité du travail de notre rapporteure. Les raisons de notre opposition sont simples. Tout d'abord, l'article 7 ne modifie pas la catégorie des personnes autorisées à présenter une offre de reprise. Il ne porte que sur l'auteur de la requête qui, depuis le 20 mai et jusqu'au 31 décembre, peut être formée non plus seulement par le ministère public, mais également par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Par ailleurs, les garanties prévues pour la mise en oeuvre d'une telle procédure restent les mêmes : le tribunal doit statuer sur la cession aux dirigeants de l'entreprise en rendant un jugement spécialement motivé, mais si la requête est formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire- ce que prévoit l'ordonnance -, alors les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, dont le recours éventuel contre le jugement est suspensif. collègues, que l'ordonnance assortit cet assouplissement de garanties supplémentaires. Ensuite, et contrairement à ce que laisse entendre notre collègue, les reprises ne bénéficient pas toujours aux dirigeants de l'entreprise. Je pense notamment à l'entreprise Camaïeu- citée par plusieurs orateurs

Madame la ministre, afin de nous rassurer, vous avez porté à notre connaissance le nombre d'offres de dirigeants effectuées sous ce régime qui ont été choisies par les tribunaux. Je vous en remercie. Enfin, mon dernier argument a trait au terme de cette disposition. L'article 10 de l'ordonnance du 20 mai 2020 prévoit qu'elle prenne fin au 31 décembre 2020.

si l'on poursuivait la navette, ce texte ne serait définitivement adopté qu'après le terme de l'application de la disposition qu'il vise à abroger. L'enjeu majeur qu'est la majeur qu'est la préservation de l'emploi dans la période actuelle implique des mesures concrètes, dont celle-ci, et une réflexion de fond, plutôt que la mobilisation de l'ordre du jour pour l'examen d'un texte qui sera en tout état de cause caduc avant de connaître le sort qui lui est définitivement réservé. La mesure contestée, salvatrice pour nombre d'entreprises, est assortie de garanties essentielles et limitée dans le temps. Aussi, le groupe RDPI ne votera pas cette proposition de loi.

L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence. » Comme parlementaires, l'établissement de ces « principes féconds » doit nous guider, que nous devons sans cesse nous interroger sur l'applicabilité des lois que nous votons. Cette exigence nous oblige devant chaque texte de loi qui nous est présenté. ces dernières années, à la procédure accélérée, le temps législatif reste un temps long. Aussi, si nous votions ce texte, il ne fait aucun doute que son adoption définitive aurait lieu après le 31 décembre 2020, et donc après qu'aura cessé l'application du dispositif qu'il vient abroger. Malgré cela,

Pour en venir au fond, le texte prévoit de mettre fin à la possibilité, ouverte par l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020, dans le contexte de crise que nous connaissons, pour un dirigeant d'entreprise de déposer une offre de rachat après avoir organisé le dépôt de bilan Le droit commun l'interdit pour plusieurs raisons. D'abord, dans un souci de moralité des affaires, il s'agit de ne pas permettre à un dirigeant d'organiser la faillite de son entreprise avant de la reprendre par la suite, délestée de ses dettes.

à prévenir les éventuelles conséquences sur l'emploi, mais aussi à soutenir les dirigeants d'entreprise qui ne sont en aucun cas responsables du contexte économique et de ses conséquences sur leurs carnets de commandes.

Aux exigences du droit commun, prévoyant que le jugement sera rendu après avis des contrôleurs, s'ajoute la présence obligatoire du ministère public à l'audience, qui peut présenter ses observations et même interjeter appel.

Néanmoins, l'exception permise par cette ordonnance doit en rester une, afin de protéger les salariés et les créanciers. Face à la poursuite de la crise sanitaire et économique, il nous faut nous interroger sur les réponses que nous souhaitons apporter à ces situations de cession, qui perdureront après le 31 décembre La mission d'information sur les outils juridiques de traitement des difficultés des entreprises nous aidera, je l'espère, à y voir plus clair et à apporter des solutions permettant de lutter contre les dérives observées.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quelques jours après le premier déconfinement, la ministre du travail d'alors, Muriel Pénicaud, a pris une série d'ordonnances,

du travail ou sur la consultation des comités sociaux et économiques. Celle du 20 mai dernier, qui nous intéresse aujourd'hui, ouvre la possibilité, pour le dirigeant d'une entreprise, de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan. du code de commerce interdisait à un dirigeant, ainsi qu'à ses parents ou alliés, de formuler une offre de reprise de sa propre entreprise dans le cadre d'un plan de cession, et ce dans un souci de moralisation des affaires, afin d'éviter les conflits d'intérêts et les fraudes, même s'il existait déjà des dérogations quand l'intérêt général le commandait. Le code de commerce, comme de nombreux éléments procéduraux en cas de faillite, a été pensé pour protéger les créanciers. Il s'agit d'éviter que le débiteur ou les dirigeants ne conservent directement ou indirectement des actifs de l'entreprise, alors même qu'ils se débarrasseraient du passif. C'est donc une protection pour l'ensemble des créanciers, entreprises et sous-traitants, mais aussi pour l'État. Il s'agit également d'empêcher la fraude à l'assurance, le non-paiement

Bien évidemment, on nous a dit : « C'est pour les entreprises qui sont en difficulté à cause de la covid. Nous serons vigilants quant aux effets d'aubaine, et le tribunal et le ministère public seront intraitables, afin que ce ne soit pas l'occasion d'effacer des dettes et de réduire les effectifs C'est évidemment raté, car de nombreuses entreprises qui ont fait appel à cette procédure avaient déjà des dettes fiscales et sociales et des plans sociaux dans les cartons avant même la crise de la covid. Les exemples sont nombreux

propriété de la famille Mulliez, dont la fortune, classée sixième de France, est évaluée à 26 milliards d'euros. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire le 13 mai 2020 et n'a pas présenté de plan de redressement viable. En conséquence, le tribunal de commerce de Marseille a validé, le 14 septembre dernier,

-, a finalement été rachetée par les mêmes propriétaires ! Comment peut-on encore nier que ce procédé de dépôt de bilan-rachat, sans garde-fou ni contrepartie, a créé un réel effet d'aubaine pour certains dirigeants, et surtout pour certains grands groupes ?

est légèrement différente. Dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la procédure est longue et les négociations avec les représentants syndicaux font que les congés de reclassement, de mobilité, les primes légales et supralégales, ou encore les plans de départ volontaire, bien mal nommés, sont plus favorables aux salariés

s'inscrivent dans le droit commun. En effet, cette ordonnance doit prendre fin le 31 décembre prochain, mais la commission des lois propose de la proroger au-delà, voire de l'inscrire dans le droit commun. Pour nous, cela est inacceptable ! Nous voterons donc

mes chers collègues, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà en peu de mots les raisons qui ont présidé à l'adoption de l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui nous occupe ce matin. En effet, ce dispositif est né de la crise et ne saurait, à ce stade, lui survivre. Entrée en vigueur alors que la France sortait à peine de son premier confinement, l'ordonnance en question répondait à l'urgence de soutenir nos entreprises les plus en difficulté. Elle complétait celle du 27 mars 2020 afin de mieux prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et de faciliter ainsi la reprise de l'activité. Souvenons-nous de notre sidération collective face à la situation inédite que nous vivions alors et qui se poursuit. Souvenons-nous des craintes et des incertitudes quant au redémarrage tant attendu et des espoirs timides de reprise. Souvenons-nous qu'il nous fallait être dans l'action pour éviter un effondrement de l'économie française. C'est dans ce contexte que l'article 7 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a été rédigé. Cette mesure a donc assoupli, jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure permettant aux dirigeants d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ou à leurs parents ou alliés, de présenter une offre d'achat partiel ou total de l'entreprise. Néanmoins, l'objet de la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui n'est autre que l'abrogation de cet article 7. Alors que le temps législatif ne s'inscrit pas toujours dans le temps très court, nous pouvons légitimement nous étonner d'un tel texte, conscients de cette échéance. Les auteurs de la proposition de loi arguent que certains chefs d'entreprise auraient profité de l'effet d'aubaine qu'offrait cet assouplissement de la procédure de reprise. Je ne peux que déplorer les quelques dérives qui sont très marginales. Ainsi s'explique, sans doute, la volonté de supprimer le dispositif de l'article 7, alors même que la crise couve toujours. Nous en mesurons les conséquences quotidiennes dans nos territoires. Cependant, peut-être que les circonstances ont obscurci les jugements ... Je n'ose croire qu'il s'agisse de voir dans tous les chefs d'entreprise des personnes sans scrupules, alors qu'ils sont les forces vives de notre économie. Plutôt que de succomber à l'émotion ou à l'idéologie, engageons un débat constructif afin de nous approcher, le plus possible, de la réalité des faits. Deux étapes se distinguent, à mon sens, en vue de suivre cette démarche. La première consiste à rappeler les motifs qui justifient l'assouplissement prévu par l'ordonnance du 20 mai 2020. Deux raisons conjoncturelles ont été retenues par le ministère de la justice

La seconde consiste à évaluer la nature du dispositif et sa mise en oeuvre. Concernant sa nature, le dispositif est d'ordre procédural : il permet au débiteur ou à 1'administrateur de former lui-même une requête en vue d'une offre de rachat, sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte. Il reste pour le moins très encadré. Outre que le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs comme le droit commun l'exige, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire. Ce dernier peut présenter, à cette occasion, ses observations et, le cas échéant, interjeter appel. Concernant la mise en oeuvre du dispositif, un examen attentif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont fait un usage prudent de la possibilité qu'il offre. Il a été le plus souvent utilisé avec l'assentiment des organes de la procédure, des salariés et du parquet, toujours en prenant en compte les spécificités de chacun des cas, et avec parcimonie. Il faut aussi rappeler que la majorité des dirigeants sont honnêtes ! Ils n'ont aucun plaisir à venir déposer le bilan de leur entreprise au greffe du tribunal de commerce, parce qu'une page de leur vie se tourne. Certains y voient même un déshonneur et garderont dans leur mémoire cet instant. En conclusion, les deux étapes d'évaluation du dispositif d'assouplissement en montrent toute la cohérence : l'idée à l'origine du dispositif est légitime et sa mise en application demeure prudente et efficace. le sort du tissu productif français, notamment des petites et moyennes entreprises qui font la richesse et le dynamisme de nos territoires, sera suspendu à ce type de mesure de soutien. J'ai une pensée pour nos restaurateurs et tous ces chefs d'entreprise qui ne peuvent toujours pas exercer leur activité à cause du maintien des mesures sanitaires. Je suis pleinement en accord avec les conclusions du rapport de la commission des lois, dont je salue le sérieux, sur une éventuelle prorogation, voire une pérennisation du dispositif. Enfin, permettez-moi de formuler un voeu, celui que le Gouvernement use de toutes les possibilités offertes par notre droit pour sauver les entreprises viables, mais fragilisées par la crise, et préserver ainsi des milliers d'emplois. Il faut conclure. Si l'État a pris des mesures indispensables pour limiter l'impact économique de la crise sanitaire, lesquelles ont d'ailleurs donné des résultats, il faut permettre

je peux aisément comprendre l'indignation de nos concitoyens lorsque les médias ont annoncé qu'il était désormais possible pour le dirigeant d'une entreprise ayant organisé son dépôt de bilan de faire une offre de rachat de sa propre entreprise.

dans des conditions strictes et contrôlées par un juge. Ainsi, il est habituellement prévu que le ministère public demande que le rachat soit autorisé, et même lorsque cette faculté est employée, rien ne garantit que le juge y ouvre droit. Cette possibilité, qui est par ailleurs très peu utilisée, est avantageuse lorsqu'il n'existe pas d'offre de rachat ou lorsque les offres sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, le maintien de l'activité et la préservation des emplois. En outre, ni la procédure de sauvegarde, ni la liquidation judiciaire, ni la cession, qui peuvent déboucher sur un rachat, ne permettent de contourner les procédures, et les règles afférentes aux licenciements économiques restent de mise si des réductions d'emplois doivent avoir lieu. Il s'agit donc d'une fausse polémique, résultant d'une désinformation, d'une méconnaissance du droit applicable, mais aussi de la diabolisation des chefs d'entreprise, lesquels chercheraient forcément à contourner la loi et à nuire à leurs employés.

J'estime naturel que le Gouvernement ait assoupli la procédure et supprimé jusqu'au 31 décembre 2020 la nécessité pour le ministère public de former une requête pour que le rachat par le dirigeant de l'entreprise puisse avoir lieu.

Devrions-nous laisser les chefs d'entreprise française tout perdre, au risque que leurs entreprises soient rachetées par des investisseurs étrangers ou, pis, qu'elles ne puissent être vendues et que tous leurs employés soient licenciés et viennent gonfler les chiffres du chômage, lesquels ne cessent de grimper ? Je suis bien conscient que cette proposition de loi a été déposée dans le but de protéger les salariés des licenciements. Cependant, mes chers collègues, nous devons garder à l'esprit que cette protection n'est possible que si nous aidons également les entreprises.

consistant à ne plus rendre la requête du ministère public obligatoire prendra fin au 31 décembre 2020. Passée cette date, la procédure habituelle reprendra. Le rachat par le dirigeant restera possible, comme cela est le cas depuis plusieurs années, mais dans des conditions plus strictes que celles qui ont pu avoir cours ces derniers mois. Il ne me semble donc pas nécessaire, à quelques jours de l'échéance de ce dispositif, de l'abroger, pas plus qu'il ne semble utile de le prolonger. Nous avons pour habitude de retravailler le droit, de l'améliorer, c'est l'un de nos rôles en tant que parlementaires. n'oublions pas que le droit est souvent bien fait et qu'il n'est pas toujours nécessaire de le modifier. Faisons confiance aux juges pour l'appliquer correctement, pour faire preuve de prudence, mais aussi de justesse, ce qu'ils ont d'ailleurs fait à plusieurs reprises ces derniers mois lorsque des propositions de rachat ont été faites par le dirigeant de l'entreprise en vente. La commission des lois a très justement remarqué dans son rapport que le droit applicable est efficace et que les modalités prévues en matière de rachats d'entreprises sont mieux connues des dirigeants, mais aussi des tribunaux, sensibilisés à la nécessité d'être souples en cette période.

chers collègues, je salue tout d'abord l'initiative de Mme Sophie Taillé-Polian et de ses collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires,

le texte ne devrait pas prospérer outre mesure. Sur le fond, la procédure de rétablissement professionnel doit permettre à des débiteurs, personnes physiques, de bénéficier d'un effacement de leurs dettes, tout en poursuivant leur activité. Il s'agit d'une procédure simplifiée, soumise à des conditions tenant notamment au montant de l'actif déclaré par le débiteur. Il est important de rappeler que le Gouvernement a souhaité étendre la possibilité pour les petits débiteurs d'utiliser cette procédure en rehaussant la valeur de l'actif en deçà duquel le débiteur est éligible à cette procédure. C'est notamment ce que prévoit l'article 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020. Cette mesure, favorable à l'utilisation de la procédure de rétablissement professionnel, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

On peut craindre que certains dirigeants, dont le comportement appellerait d'éventuelles sanctions, puissent contourner les règles applicables en demandant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel pour effacer les dettes de leur entreprise sans contrôle suffisant. Ces quelques éléments de réponse permettront de nourrir une réflexion plus générale sur l'amélioration des procédures des tribunaux de commerce au service des entreprises en difficulté.

Notre assemblée s'est d'ailleurs saisie du problème une délégation chargée du travail parlementaire, qui s'est vue logiquement confier la mission de contrôle et de suivi des ordonnances. Je trouve regrettable que les sénateurs doivent,

Je vous rappelle que la commission est défavorable à cet article, qui vise à ratifier l'intégralité de l'ordonnance du 20 mai 2020. Le Parlement ne saurait ratifier cette ordonnance sans un examen plus approfondi qui dépasse le cadre de cette proposition de loi. L'ordonnance du 20 mai 2020 comprend de nombreuses dispositions, dont certaines ont appelé des réserves de la part de nos collègues François-Noël Buffet et Patrick Kanner, rapporteurs de la mission de suivi de la commission des lois sur la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire.

est aujourd'hui discutée par votre Haute Assemblée. Cette proposition de loi nourrit une ambition que nous avons tous en partage et qui figure depuis 2008 en toutes lettres dans notre Constitution, à l'article 75-1 qui dispose : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. au patrimoine de la France. » Par ces mots, ce sont les attaches et les cultures de nos concitoyens qui sont reconnues. Par ces mots, ce sont les richesses des pays et des langues qui ont été et sont pleinement considérées comme parties prenantes de l'identité de chacun d'entre nous. Comme la philosophe Simone Weil l'écrivait, nous savons que « l'enracinement est peut-être [notre] besoin le plus important et le plus méconnu. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines.

n'est non seulement pas incompatible, mais se nourrit des appartenances locales qui sont évidemment aussi la sève de notre beau pays. Aucune société ne se projette avec confiance dans l'avenir sans de tels attachements. Tel est d'ailleurs le projet même de notre école : donner à chaque enfant des racines, par la transmission des savoirs des siècles passés, et lui donner des ailes, par l'accès aux connaissances les plus modernes. C'est bien pourquoi, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis un partisan de l'enseignement des langues régionales : il est pour moi évident que les langues de nos régions figurent parmi les trésors culturels que compte notre pays ; j'ai également la conviction qu'elles contribuent à l'accomplissement intellectuel et sensible d'un être humain.

L'éducation nationale s'est pleinement saisie de cette richesse pour la proposer à nos élèves et la faire vivre. C'est pourquoi l'on ne doit jamais caricaturer ni notre pays ni notre système éducatif comme étant hostile aux langues régionales : ce n'est pas vrai

discipline en 2019. Tous ces professeurs permettent aujourd'hui à 170 000 de nos élèves d'apprendre une langue vivante régionale. Chaque jour, nous nous attachons à faire progresser ce chiffre en proposant un parcours cohérent depuis l'école jusqu'au lycée. J'en veux pour preuve la place ménagée aux langues régionales dans la réforme du lycée général et technologique. Aujourd'hui, avec le nouveau lycée, un élève peut choisir de suivre un enseignement de langue et de culture régionales

mais aussi comme langue vivante C, dans le cadre d'un enseignement optionnel, ce qui est le cas pour 3 389 élèves ; et, enfin, comme enseignement de spécialité sur le cycle terminal, avec des programmes riches et ambitieux adossés à des coefficients importants- 16 sur 100 au baccalauréat 134 élèves de première sont concernés, et nous attendons les chiffres pour la terminale. Nous avons donc démultiplié les possibilités d'apprendre une langue régionale au lycée, en maintenant les mêmes volumes horaires et, surtout, en proposant, avec les nouveaux enseignements de spécialité, des horaires importants qui permettent aux élèves de découvrir de manière approfondie les caractéristiques, tant des langues que des cultures régionales. J'ai entendu les critiques sur les difficultés que rencontreraient certains lycéens pour suivre un enseignement en langue régionale. Assurément, nous pouvons çà et là améliorer l'offre et le maillage, et je continuerai à m'y employer. Pour autant, sachons tirer le bon diagnostic de la situation actuelle

Ils disposeront ainsi d'une offre de formation de qualité, qui pourra s'appuyer sur un accompagnement dans leur établissement par un professeur aux compétences reconnues. Nous pouvons également progresser dans d'autres domaines. Je pense à la formation initiale, et en particulier à des modules spécifiques pour l'enseignement du bilinguisme. Notre action n'est pas isolée : elle est pleinement concertée avec les acteurs et les défenseurs des langues régionales, qui siègent dans les conseils académiques des langues régionales, et qui font vivre ces langues au sein des offices publics de langue régionale. Ces différents éléments, mesdames, messieurs les sénateurs, n'en sont que quelques-uns parmi d'autres que je pourrai développer tout à l'heure. Ils vous auront cependant permis de mesurer l'engagement de notre ministère pour la promotion des langues régionales. Alors, pourquoi avoir supprimé les articles 3 à 7 de cette proposition de loi, qui portaient justement sur l'enseignement des langues régionales ? J'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale le 14 février dernier, et je le redis aujourd'hui : les différents sujets traités dans ces articles ont déjà été discutés voilà plus d'un an dans le cadre de la loi pour une école de la confiance. Le Parlement a donc déjà tranché. Sur d'autres aspects, plusieurs articles et amendements étaient de pure forme. Ils étaient la plupart du temps déjà satisfaits.

en ce domaine, l'exigence d'équilibre s'impose et, en matière d'enseignement, cet équilibre doit se manifester à travers le respect des deux langues enseignées, qui peut aller jusqu'à la parité horaire dans le cadre de l'enseignement bilingue. L'enseignement des langues régionales est un aboutissement et l'expression de notre idéal français, celui que nous avons construit au travers de notre histoire, et qui consiste précisément en une juste articulation entre la Nation et le pays, entre l'ambition de partager une même langue, de porter un message et des valeurs qui nous élèvent en tant que Français, et la reconnaissance bien légitime de nos attaches. Le sujet n'est pas nouveau, nous le savons : il a déjà été éclairé par un avis du Conseil d'État en 2002. Je m'y tiendrai scrupuleusement, et je m'y tiendrai d'autant plus que je suis convaincu que les premières années d'apprentissage du français sont absolument fondamentales : c'est cette même conviction qui m'a conduit à défendre l'abaissement de l'instruction obligatoire à trois ans. Aussi, l'expérimentation d'un enseignement immersif doit rester l'exception, une exception issue d'une demande légitime et soumise à un cadre, un protocole, une régulation et une durée déterminés. donc pas d'une opposition de principe, mais de faire valoir notre grande priorité, qui est aussi un devoir à l'égard des enfants, à savoir la qualité de l'enseignement du français pour tous nos élèves. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, j'aborderai la proposition de loi qui est au centre de nos échanges aujourd'hui avec une ambition et des exigences chevillées au corps : l'ambition de faire mieux pour la promotion et l'enseignement des langues régionales, l'exigence du discernement et de la mesure, afin de garder toujours à l'esprit les efforts déjà déployés et le nécessaire respect de nos différents engagements et, enfin, l'intérêt des élèves et le respect du cadre juridique, qui constituent nos boussoles.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Elles constituent une richesse culturelle, patrimoniale et linguistique pour notre pays. Le ministère de la culture en dénombre une vingtaine en France métropolitaine, et plus d'une cinquantaine dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, ces langues sont aujourd'hui menacées. Selon le classement de l'Unesco, les langues de France sont soit vulnérables, soit en danger, soit sérieusement en danger. Un premier constat peut être dressé : nous connaissons très mal le nombre de locuteurs de langues régionales. La dernière enquête nationale date du recensement de 1999. L'Insee avait alors évalué à 5,5 millions le nombre de personnes déclarant que leurs parents leur parlaient dans une langue régionale. C'était il y a plus de vingt ans, soit une génération. Quelle est la pratique de ces langues aujourd'hui ? Certes, des collectivités territoriales, comme la région Bretagne, chère à Sylvie Robert, Ronan Dantec et bien d'autres, ou des associations ont pris l'initiative de lancer des études sur le nombre de locuteurs. Par exemple, l'occitan, dans l'ensemble de ses variantes, serait parlé par un million de locuteurs. Mais il nous manque une vision nationale actualisée. Comment construire Comment construire une politique ambitieuse de promotion des langues régionales si nous ne disposons pas d'une connaissance précise du nombre de locuteurs et de la situation de chaque langue ? Monsieur le ministre, il me semble important qu'une nouvelle enquête nationale Cependant, même en l'absence de données précises, chacun s'accorde à dire que la pratique des langues régionales est en baisse. Si la pratique des langues régionales ultramarines résiste bien, tout comme celle du breton et du basque, la pratique des autres langues connaît une forte diminution. À titre d'exemple, en l'espace de vingt ans, le nombre de locuteurs du flamand occidental a été divisé par deux, en raison du manque de soutien politique. Et encore, cette langue régionale a la chance d'être transfrontalière et de bénéficier du dynamisme linguistique en Belgique. Mes chers collègues, prenons conscience de la situation d'autres langues régionales qui ne sont pratiquement plus transmises dans le cercle familial, qui ne peuvent pas s'appuyer sur un vivier linguistique transfrontalier et qui ne bénéficient pas d'un volontarisme politique pour les promouvoir et les défendre. Deuxième constat : la valorisation et la promotion des langues régionales passent par leur utilisation et leur transmission. Le service public France Télévision et Radio France propose des programmes bilingues ou en langue régionale. Peut-être pourraient-ils être plus nombreux

Aussi la commission a-t-elle regretté qu'un texte visant la promotion des langues régionales nous soit transmis amputé de ses principales dispositions relatives à l'enseignement des langues régionales. C'est pourquoi la commission a donné un avis favorable à plusieurs amendements tendant à encourager et à faciliter leur enseignement. Nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de nous emparer de ce sujet à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de Paul Molac. D'ailleurs, la thématique des langues régionales avait animé le Sénat lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Notre collègue Max Brisson, dont chacun connaît l'attachement à la langue basque, et qui était rapporteur de ce texte, peut en témoigner. Monsieur le ministre, plusieurs intervenants nous ont par ailleurs alertés sur les conséquences de la réforme du baccalauréat pour l'enseignement des langues régionales. Les difficultés relèvent principalement de l'échelon infralégislatif. Votre ministère a donc la possibilité d'agir rapidement pour promouvoir les langues régionales. Je pense tout d'abord à la comptabilisation des notes des épreuves de langue régionale pour le baccalauréat. Serait-il possible que le mode de calcul appliqué au latin et du grec ancien le soit également aux langues régionales ? Ces deux langues anciennes sont les seules options pour lesquelles le bonus des points au-dessus de la moyenne est maintenu. De plus, ces points sont affectés d'un coefficient de 3. Par ailleurs, je suis avec intérêt la réflexion en cours pour développer, le CNED, un enseignement à distance des langues régionales. Un tel dispositif permettrait à un élève de présenter cette matière au baccalauréat, même si l'enseignement n'est pas proposé dans son établissement ou s'il n'a pas pu le suivre. Il pourrait également intéresser un public plus large souhaitant se former à une langue régionale. J'espère que cette démarche pourra aboutir. J'en viens enfin à mon quatrième et par méconnaissance, mais aussi par manque de volontarisme politique, les nombreux outils de promotion et de valorisation des langues régionales ne sont pas suffisamment exploités. Aussi, ce texte vise à préciser l'articulation entre le français et le recours aux langues régionales. Il a également pour objet de lever les ambiguïtés sur l'utilisation des langues régionales dans l'espace public et pour les actes d'état civil. Le Conseil constitutionnel l'a clairement indiqué dans sa décision relative à l'emploi de la langue française de 1994 : l'usage des traductions, notamment en langue régionale, est possible dès lors que l'utilisation de la langue française est assurée. Néanmoins, dans les territoires, on constate de nombreuses interrogations sur la possibilité de recourir à des traductions en langue régionale. Il me paraît important d'apporter une réponse juridique claire à tous les promoteurs de ces langues. Monsieur Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est désormais urgent d'agir pour promouvoir les langues régionales. Sans volontarisme politique fort, la plupart de ces langues auront disparu dans quelques dizaines d'années ou seront vues comme des curiosités historiques. Cette proposition de loi doit leur permettre de rester un patrimoine vivant de notre pays. La parole

cette proposition de loi est une nouvelle occasion d'opposer les jacobins centralisateurs aux girondins défenseurs de la diversité culturelle et linguistique. Le principe d'une République une et indivisible s'applique jusque sur le plan linguistique. Pourtant le bilinguisme français-langues régionales est une vraie richesse au niveau intellectuel et éducatif. Les jeunes Français ne sont pas les plus brillants en langues étrangères, mais un jeune bilingue français-langues régionales aura beaucoup plus de facilité pour apprendre plus vite et mieux une troisième, voire une quatrième langue. À l'heure de l'Europe des régions et de la mondialisation, le jacobinisme est un réflexe de peur et de repli sur soi. La rupture avec ce jacobinisme a été amorcée à la fin des années 1970, mais c'est surtout l'engagement des socialistes qui a permis de faire entrer cette question dans le débat politique. De nombreuses avancées ont pu voir le jour, notamment sous la présidence

en 2013, la participation financière dans la loi NOTRe, la proposition de loi des députés socialistes de 2016, cosignée par le député-rapporteur Paul Molac,

Parce qu'une langue qui meurt entraîne la perte irrémédiable de la connaissance et d'une part de notre identité, dans le domaine culturel, historique et environnemental. Chaque langue témoigne de l'expérience humaine. La maîtrise des langues apporte une réponse aux questions fondamentales de demain. Or une évolution est en cours, lente et insidieuse. L'anglais et les anglicismes envahissent de plus en plus la langue française. Certains linguistes y voient, au mieux une perte des repères culturels, au pire une rampante victoire idéologique du libéralisme anglo-saxon. Défendre nos langues régionales, c'est donc défendre nos valeurs, comme héritage direct de notre histoire. Les langues régionales consacrent la pluralité et la diversité de nos territoires. La proposition de loi soumise à notre examen aujourd'hui est importante : elle institue la reconnaissance de l'intérêt patrimonial des différentes langues régionales, qui bénéficieront désormais d'actions de conservation et de promotion. Une langue, c'est une perception du monde, une école de pensée, une culture. Une langue, c'est une façon de vivre, de percevoir et de transmettre le monde. C'est le vecteur d'un héritage, d'une histoire passée, mais aussi celui de la transmission des conditions d'un renouveau dans notre conception de la Nation. Les langues régionales sont une partie intégrante de notre patrimoine et leur richesse culturelle construit notre identité. Toutes les langues, quelles qu'elles soient, offrent un témoignage unique de notre génie culturel. Afin de préserver la diversité linguistique de notre pays, l'usage et la présence au quotidien de nos langues régionales sont cruciaux. Si les domaines de l'état civil et de l'espace public abordés dans cette proposition de loi en sont deux composantes essentielles, le champ de l'éducation ne doit pas être négligé. Les amendements qui ont pris corps lors de nos échanges en commission, concernant l'extension du dispositif appliqué en Corse et la suppression du caractère volontaire de la contribution financière, ont été repris. Notre groupe les fait siens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, charmes de la France métropolitaine et de nos outre-mer, nos langues régionales sont les accents variés de notre langue nationale. Elles sont les rivières qui viennent se jeter dans l'océan français. Les articles 3 et 7, à l'origine de cette proposition de loi en faveur de l'enseignement bilingue, étaient les plus engageants pour l'État. Ils ont disparu depuis. Toutefois, il existe déjà de nombreuses dispositions dans la loi qui vont dans ce sens. Par ailleurs, nous constatons que le niveau de l'enseignement de la langue française est en baisse constante. Il est urgent que nos enfants apprennent le français autrement que par la méthode globale, qu'ils écrivent autrement que par les SMS et qu'ils ne soient plus soumis au verbiage abrutissant de musiques « urbaines » qui riment avec « haine », haine de tout ce qui fait la France, y compris sa langue. Faite de subtilités, celle-ci est l'expression de notre culture commune, l'actrice ô combien vivante et vivace de notre histoire. La langue dit qui l'on est, d'où l'on vient. Elle est un élément essentiel de la cohésion nationale. Clovis, qui étendit ses États de la Loire jusqu'au Rhin, parlait germanique et ce fut la rencontre avec le latin des Gallo-Romains qui donna naissance à la langue francique, jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, par laquelle le roi François I imposa le français pour la rédaction des actes légaux et notariés. Mais il faut attendre la fin du XIX siècle pour qu'il devienne la langue de tous les Français. Écouter la langue française, c'est entendre l'histoire de France ! Parler français, c'est rendre hommage et faire honneur à ceux qui ont fait notre pays ! Notre patrimoine linguistique est varié, il faut le valoriser. Il faut que nous soyons capables de valoriser également l'enseignement des langues latines et grecques dans nos écoles, car elles sont le coeur sémantique de notre langue. Mais c'est la même République qui a fait interdire le provençal dans les cours d'école pour imposer l'unité nationale, qui veut désormais imposer l'enseignement de la langue arabe pour mieux valoriser l'autre. la haine de soi va jusqu'à l'ethno-masochisme ... Menteur ! Le français s'enrichit de la diversité linguistique de ses territoires. Les langues régionales rappellent à chaque région leurs réalités historiques, géographiques et identitaires. Un Provençal n'est pas un Breton, qui n'est pas un Corse, qui lui-même n'est pas un Martiniquais. Si tous sont fiers de leur petite patrie, tous s'unissent en admettant qu'elle ne saurait être au-dessus de la grande. Félix Gras, disciple de Frédéric Mistral, nous rappelle cette nécessaire hiérarchie du sentiment d'appartenance : « J'aime mon village plus que ton village, j'aime ma Provence plus que ta province, j'aime la France plus que tout ! » Il est là, le génie français Accordons dès lors à nos territoires, à nos communes la possibilité de promouvoir nos langues régionales. Dans le fracas de l'uniformisation imposée par la mondialisation et face à la montée du communautarisme sous perfusion migratoire, pour que le français ne soit pas une langue morte, il faut que vivent nos langues régionales ! Il y va de l'intérêt culturel local et de notre patrimoine national ! Pour conclure, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette fin d'année 2020, comme nous le disons encore au Roudelet Felibren et au groupe Saint Éloi de Casteou Gombert

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chère Monique de Marco- dont je voudrais saluer la qualité du travail -, mes chers collègues, ni la France ni la République n'ont eu de rapports faciles avec les langues de nos territoires qualifiées de « régionales ». Celles-ci furent longtemps le symbole de la France restée celle du cheval de trait, archaïque, voire réactionnaire. Beaucoup de nos langues, appelées alors avec plus ou moins de mépris « patois », ne résistèrent pas au rouleau compresseur de la modernité. L'école a contribué à ce recul. Mais l'urbanisation et la télévision jouèrent finalement, à partir des années 1950 et 1960, un rôle au moins tout aussi grand dans la rupture de la transmission familiale. Pour autant, nous ne sommes plus en 1950. Nos langues, au moins là où elles ont survécu, si elles ne sont pas autant parlées dans les rues de nos villages et encore moins de nos villes, le sont désormais à l'école, où elles furent longtemps interdites inversion de situation, caractérisée par un recul de nos langues dans la société, mais par une irruption salvatrice à l'école. Devons-nous le relever et le saluer ? Oui, monsieur le ministre Devons-nous nous en contenter ? Non, monsieur le ministre ! Car c'est sur l'école que reposent, désormais, la préservation et le développement de nos langues. C'est un renversement historique Or si l'institution scolaire a fait des efforts, elle n'a jamais intégré la notion de politique linguistique et son objectif final, la production de locuteurs complets, sachant vivre et travailler dans leur langue. Dans nos territoires, l'éducation nationale a trop souvent un train de retard, car elle n'intègre pas le réveil des langues, la demande sociale et l'appétence des jeunes générations pour ce qui est un élément du réveil des territoires. Au Pays basque par exemple- je le dis sous le contrôle de Frédérique Espagnac nous avons compris depuis longtemps que les territoires sans identité étaient des territoires sans projet. La langue appartient certes au patrimoine, mais elle est d'abord un facteur d'attractivité, et finalement, loin d'une approche muséographique et nostalgique, elle s'inscrit pour nous comme un facteur de modernité. Elle est aussi, loin des fantasmes jacobins, un vecteur d'intégration, de solidarité et de préservation du tissu social, dans un pays où il se délite si souvent. Dans ces conditions, s'il faut féliciter Paul Molac pour sa proposition de loi- et je tiens à saluer sa présence dans nos tribunes -, il faut regretter que l'Assemblée nationale ait exfiltré tous les articles du texte qui concernaient l'enseignement, comme s'il pouvait y avoir une politique en faveur des langues régionales sans renouveler, fortifier, conforter la transmission l'école. Depuis la loi Deixonne, ce n'est en effet que par les marges que l'éducation nationale aborde le sujet, en annexe de lois majeures

française, pourtant voulue pour lutter contre l', fut rarement utilisée face à la percée de l'impérium anglo-américain, mais très souvent contre les langues de France. services de l'éducation nationale (Dasen) se draper dans cette loi de 1994, trahissant la volonté du législateur à tel point que mon ami Alain Lamassoure m'indiquait un jour que, s'il avait su comment cette loi serait instrumentalisée, il ne s'y serait pas associé. Je conclurai en disant mon soutien à cette proposition de loi, qui rappelle l'État à ses obligations : préservation de ce patrimoine immatériel, sécurisation juridique de la présence des langues régionales dans les espaces publics, utilisation des signes diacritiques, cadrage de la loi Toubon. Il faudra aussi parler de l'école, et ce sera l'objet des amendements que nous défendrons. Nos langues de France sont une richesse. Le pays qui prône, ou du moins prônait, l'exception culturelle ne peut laisser dépérir ce trésor inestimable. Le développement durable, c'est la transmission aux générations de demain d'un capital naturel et humain. Il est de la responsabilité de notre génération d'assurer cette transmission, pour les générations futures. Dans certains territoires de France, ce matin,

nous regardent et attendent que nous soyons à la hauteur des générations qui nous ont précédés et qui aimèrent et parlèrent leur langue maternelle. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la France est un État historiquement multilingue. On y trouve de nombreux locuteurs de langues romanes, comme le français, l'occitan, le catalan, le corse, le le catalan, le corse, le francoprovençal, mais également de langues germaniques, comme l'alsacien, le flamand occidental et le ou encore du basque et du breton- pour ne parler que de la France métropolitaine. Le texte de notre collègue Paul Molac, présent dans nos tribunes, tend à considérer toute la pluralité des langues dans notre pays. Il importe de changer le regard que l'on pose traditionnellement sur les langues régionales. Ces langues sont au français ce que nos territoires sont à la France. J'aimerais vous citer un- excusez l'expression ! -sans équivoque du président de la République, en date du 21 juin 2018 : « Les langues régionales jouent leur rôle dans l'enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. Aujourd'hui, après plus de deux années, nous débattons d'une proposition de loi, dont l'un des objectifs principaux est bien d'enseigner nos langues de France. Ce texte, débattu en premier lieu à l'Assemblée nationale, a été vidé de sa substance avant d'arriver dans cet hémicycle. Nous pouvons le regretter. Toutefois, les amendements visant à redonner du corps à la proposition de loi, en rétablissant l'article 3 et en permettant le versement d'un forfait scolaire de l'enseignement bilingue, sont de bon ton et ambitionnent de donner une réalité, au sein de l'école de la République, à nos langues régionales. Nous serons nombreux à les soutenir. La défense et la promotion des langues régionales, ce n'est pas une lubie ; c'est encore moins une revendication communautariste. Il faut sortir de ce paradigme. Le coeur de cette proposition de loi est bien d'inclure les langues régionales au sein de nos institutions, afin qu'elles participent à la vie de la cité. Nos concitoyens y sont attachés. Il est important de soulever un point essentiel. Pour la réussite de tels projets, l'État doit associer les collectivités territoriales et leur laisser une marge de manoeuvre. Bien entendu, ces dernières n'ont pas attendu pour s'organiser ! Localement, on constate que de nombreux acteurs sont investis dans la défense et la promotion des langues régionales, pour l'acceptation de leurs identités. Dans les Hauts-de-France, je veux souligner le soutien actif du conseil régional, avec, notamment, la création d'un office public du flamand Nos langues régionales ont fait preuve d'une grande résilience, voire de résistance, et restent des réalités. Pourtant, il y a urgence à agir, avant qu'elles ne soient plus que des folklores destinés à mourir tôt ou tard. Bien que la Constitution érige les langues régionales au rang de patrimoine de la France, ces langues ne doivent pas être mises sous cloche ni admirées comme des vestiges du passé. Comme l'a si bien dit notre collègue Paul Molac, « une langue ne s'abîme pas quand on la parle, mais uniquement quand on ne la parle pas L'enseignement est la seule manière viable et de long terme pour protéger et promouvoir les langues régionales. Jean Jaurès, dans la du 15 octobre 1911, s'étonnait déjà qu'un enfant parlant l'occitan, avec un réflexe d'analogie et de comparaison, déchiffrât aisément le portugais, l'espagnol et même l'italien. Les langues régionales étaient pour lui un moyen d'être « en harmonie naturelle, en communication aisée avec ce vaste monde ». En somme, l'apprentissage de la langue de sa région est un avantage pour mieux se lancer dans le monde. Je tiens à rappeler que, au sein de l'Union européenne, on dénombre plus de 60 langues régionales ou minoritaires. Monsieur le ministre, avec un peu de bonne foi, ce qui se dessine dans la dernière réforme du lycée ouvre la possibilité de créer des cursus d'enseignement de certaines langues régionales. Toutefois, il faut préciser que toutes ces langues ne sont pas logées à la même enseigne. Ces disparités sont parfois vectrices de frustrations et d'incompréhension. Je pense, bien entendu et vous le savez,

À ce propos, je vous remercie, madame la rapporteure, de votre détermination. La proposition de loi que nous examinons vise à pérenniser et valoriser une partie de notre culture et de nos patrimoines. En l'espèce, ce n'est pas la panacée. Les dispositions de ce texte vont dans le sens d'une plus grande reconnaissance de nos langues régionales, des particularités de nos territoires et de leurs habitants. Cela nous permet de rappeler à quel point notre pays est beau et fort de sa pluralité. Le groupe Les Indépendants votera donc cette proposition de loi.

je suis aujourd'hui sénatrice du Finistère, mais je dois vous faire une confidence : je ne parle ni le gallo ni le breton. Parfois, je tente.

Mais, à vrai dire, je ne parle pas non plus l'alsacien, le francique-mosellan, le basque, le créole, le corse ou l'occitan, pas plus que le catalan, le wallisien et futunien ou le tahitien.

En fait, je parle le français, et l'espagnol par mes origines familiales. J'ai voulu consulter les autres membres de mon groupe sur la signification que revêtaient, pour eux, les langues régionales, et j'ai voyagé, de départements en régions, de souvenirs d'enfance en moments plus présents. Sans les parler donc, j'essaierais toutefois, dans les quelques minutes dont je dispose, de rappeler leur appartenance à notre patrimoine commun et d'en défendre l'apprentissage, puisque tel est l'objet de la proposition de loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale et dont un grand nombre d'articles a été adopté conforme par les membres de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. Je voudrais expliquer pourquoi Partons, tout d'abord, d'une définition la plus simple possible : une langue régionale est, du point de vue géographique, parlée dans une région faisant partie de l'État, plus vaste. D'un point de vue historique, elle est parlée depuis plus longtemps que le français. Partons, ensuite, d'un constat : la pratique des langues régionales, richesse linguistique de notre pays, est aujourd'hui en baisse. À ce propos, je cite le linguiste George Steiner, décédé en début d'année La mort d'une langue, fût-elle chuchotée par une infime poignée sur quelque parcelle de territoire condamné, est la mort d'un monde. Chaque jour qui passe s'amenuise le nombre de manières de dire " espoir Rappelons enfin ce qui doit être une évidence : notre attachement profond au principe d'unicité du peuple français et d'indivisibilité de la République. Ainsi peut-on lire, à l'article 2 de notre Constitution, « la langue de la République est le français ». Toutefois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, a introduit un article 75-1, nouveau, portant la mention suivante : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » C'est un équilibre à trouver, dans un cadre qu'il nous faut préserver et par l'échange. J'oserai presque dire qu'il nous faut parvenir à ce « en même temps », mais suis-je dans la bonne assemblée pour cela ? Lors de sa visite à Quimper en 2018, dix ans après la révision constitutionnelle, Emmanuel Macron avait affirmé vouloir soutenir les langues régionales.

peut très bien aller de pair avec une politique dynamique au service des langues régionales. » Je partage ce point de vue. Depuis votre arrivée, l'offre a été renforcée face à la baisse massive, au collège et au lycée, des effectifs d'élèves étudiant La loi précédemment évoquée a étendu à l'enseignement privé les dispositions relatives à la prise en charge du forfait scolaire dans le cas où un élève s'inscrit dans une école située en dehors de sa commune de résidence pour y recevoir un enseignement en langue régionale. Un amendement déposé par des parlementaires présents sur ces travées, et sensibles à ces questions, sera discuté ultérieurement, de même que sera abordée la question du conventionnement. Notons que la réforme du baccalauréat veut faire une meilleure place aux langues régionales dans les épreuves de cet examen. Mon groupe est attaché à la défense et à la reconnaissance des langues régionales comme partie de notre patrimoine immatériel. Nous sommes donc favorables, collectivement, à certaines dispositions, notamment aux articles 1 et 2. Nous sommes aussi tout à fait favorables à l'esprit de l'article 8, qui tend à renforcer la visibilité des langues régionales et leur immersion dans la vie quotidienne, gages de leur pleine transmission. Les langues et cultures régionales sont structurantes pour les territoires, pour nos régions et pour leur attractivité. Elles en traduisent l'histoire, la culture. Elles sont un lien intergénérationnel et familial. Chacun reconnaît l'intérêt du plurilinguisme pour le développement cognitif des enfants. L'ouverture à d'autres langues et cultures, qu'elles soient régionales ou étrangères, s'inscrit dans une démarche positive et ne remet pas en cause le français comme langue de la République. Surtout pas !

quelle langue parlerions-nous si la monarchie s'était installée à Toulouse ? L'occitan probablement ! Nous connaissons bien les conditions historiques de l'ancrage du français. Les monarques, de Louis XI à François I- et la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts -, puis les révolutionnaires de 1789 : tous ont convergé vers un même principe

ce n'est pas si vieux, le français n'était pas encore partout la langue usuelle. Voilà cent ans, mon grand-père était instituteur en Aveyron. Il m'a raconté comment il accueillait des élèves qui ne parlaient pas la langue française. À la ferme, on ne parlait pas le français. Parce que les langues régionales ont aussi constitué le symbole de la résistance au pouvoir central, un sentiment a longtemps perduré, une certaine méfiance à leur encontre. Aujourd'hui, nous avons heureusement passé ce cap. Il est bien acquis que la République est indivisible : ce principe constitutionnel n'interdit pas pour autant la coexistence du français avec le parler de nos territoires.

Plusieurs textes adoptés depuis la fameuse loi Deixonne de 1951 illustrent l'ouverture du législateur à la promotion des langues régionales. Face au risque de leur extinction, nous pouvons toutefois aller plus loin, comme le propose le texte de notre collègue député Paul Molac. Est-il utile de rappeler ici, au Sénat, maison des collectivités locales, combien la diversité linguistique est une richesse ? Je passerai vite sur l'impact positif du bilinguisme sur le développement cognitif des enfants. C'est une affaire de spécialistes ! Seulement par quelques mots, je dirai que les études tendent à démontrer tout le bénéfice de ce que les linguistes appellent « la conscience métalinguistique Plus simplement, comme certains orateurs l'ont rappelé, les langues régionales sont avant tout constitutives de notre patrimoine. Elles alimentent la richesse de nos territoires, leur attractivité culturelle. Aussi mon groupe est-il plutôt favorable aux deux premiers articles de ce texte, dont le dispositif renforce la protection patrimoniale des langues régionales. Si, en 2008, le législateur a intégré les langues régionales à notre Constitution, leur inscription au code du patrimoine marquerait en effet une étape supplémentaire pour leur valorisation et leur conservation. L'usage d'une langue locale répond aussi à un besoin d'affirmation identitaire, dans un monde très ouvert où la perte des repères et des racines s'accélère. Là aussi, la proposition de loi apporte une réponse : je pense, en particulier, à l'article relatif à la faculté d'utiliser les signes diacritiques dans les actes d'état civil, ainsi qu'à l'article visant à conforter la traduction en langue régionale des inscriptions publiques.

s'agissant de la participation financière des communes à la scolarisation, en prenant garde, toutefois, à ne pas fragiliser le tissu des petites écoles en milieu rural. Enfin, mes chers collègues, le texte ne l'aborde pas, mais il y a d'autres moyens pour valoriser notre patrimoine linguistique. Je pense aux médias. Cette valorisation fait ainsi partie des missions de service public de France Télévisions et Radio France.

Mes chers collègues, attentif à tout ce qui valorise la diversité des territoires, le groupe du RDSE est favorable à la proposition de loi. Nous espérons qu'elle contribuera à faire vivre toutes nos belles langues locales.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré les difficultés méthodologiques de décompte, on estime aujourd'hui qu'un peu plus de 7 % de la population en France est locutrice régionale, contre un quart il y a cent ans. Ce déclin, attribué à de nombreux facteurs, doit nous interroger. Nous devons surtout nous rappeler notre histoire. Les langues régionales ont connu, dès la Révolution française, un sort particulier. D'abord promues en 1790, car permettant une meilleure compréhension des lois et décrets, elles ont pâti dès 1794 de la politique linguistique de la Convention qui, en imposant le français partout, souhaitait construire l'unité de la Nation. Dans un pays où, à quelques centaines de mètres d'écart, on n'avait ni la même langue, ni la même monnaie, ni la même unité de mesure, c'était une nécessité. La fragile Troisième République a poursuivi cette politique d'effacement des langues régionales. Ce faisant, elle souhaitait une nouvelle fois l'union nationale et la consolidation du régime républicain face aux particularismes. Aujourd'hui, notre République s'est consolidée par l'unification de la langue et le renforcement de l'État national. La question des langues régionales doit donc se poser autrement. Il me semble qu'il faut réaffirmer qu'elles sont une richesse nationale. Elles témoignent tout à la fois de l'histoire de France et de la construction difficile de l'État : comment nous sommes passés de la féodalité à la République en passant par la monarchie centralisée ; comment un peuple divisé et cloué sur son sol a pu s'unir dans un projet commun ; comment ce dernier s'est aussi enrichi grâce à la diversité, notamment linguistique, de ses habitants. Il est loin le temps où Voltaire, voulant se rendre à Uzès, se plaignait d'avoir besoin d'un traducteur. Le français lui-même s'est enrichi des langues régionales en intégrant, au sein de son vocabulaire et de sa grammaire, des mots régionaux. Le « maquis » corse rencontrait, grâce à ce cadre commun qu'est le français, le « béret » béarnais, la « brioche » normande ou le « guignol » arpitan. Et c'est bien en intégrant, en captant ces mots que le français s'est enrichi, s'est implanté durablement et a suivi la vocation d'une langue vivante, à savoir évoluer. Cette proposition de loi revêt donc une dimension symbolique très forte, d'autant plus que la majorité de ses articles sont déjà couverts, partiellement ou totalement, par le droit en vigueur. On peut d'ailleurs le regretter. En effet, malgré les dispositifs existants, nous voyons bien les difficultés actuellement rencontrées pour pérenniser les langues régionales. Cela veut dire que la protection actuelle n'est pas assez efficace. À titre d'exemple, l'augmentation des moyens accordés à l'éducation nationale publique pour qu'elle multiplie les cursus de langues régionales et le développement des initiatives locales devient un enjeu central. L'Assemblée nationale a judicieusement supprimé une partie des dispositions de la proposition de Oui, la défense des langues régionales en tant que richesses nationales est nécessaire. Dans ce cadre, il est central que les initiatives permettant d'apprendre et de parler ces langues soient soutenues. En ce sens, les associations régionales de médiation culturelle et linguistique font un travail remarquable qu'il me faut saluer. Notre Constitution pose, en la matière, trois principes que je veux rappeler : premièrement, la République est une et indivisible, et ne saurait donc se morceler sur un modèle fédéral ; deuxièmement, sa langue est le français ; troisièmement, comme je l'ai développé plus haut, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. En l'état, cette proposition de loi trouve un juste équilibre, quoique précaire ; avec mon groupe, nous la soutiendrons. Mes chers collègues, un consensus s'est dégagé au sein de notre commission- et se dégagera probablement dans notre hémicycle -sur les enjeux de ce texte. Nous avons tous à coeur de défendre ce qui a fait la beauté de ce pays, son ancrage et sa diversité. Toutefois, certaines lignes rouges doivent être maintenues